d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je salue la présence dans notre tribune d'honneur de Mme Martine Biron, ministre des relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine du Québec. Elle est Elle est accompagnée par le président du groupe d'amitié chers collègues, la chaleur et la spontanéité de vos applaudissements attestent de la qualité de la relation que nous avons avec le Québec. Nous souhaitons à Mme la ministre la bienvenue dans notre hémicycle et un fructueux séjour en France.

Cette situation a occasionné des débats parfois vifs, souvent passionnés, s'agissant d'un problème extrêmement grave, mais aussi très complexe. Ma première question : quelle est la doctrine de notre pays ? Est-ce celle qui a été exprimée par M. le Président de la République en 2018 ou est-ce celle de la jurisprudence Toulon 2022 ? Par ailleurs, nos frontières sont essentiellement européennes. La crise migratoire touche à nos sociétés ; c'est un sujet qui constitue une affaire incandescente pour toutes nos sociétés européennes.

Nous discutons de moins en moins avec nos amis au sein de l'Europe : nous nous éloignons de l'Europe, nous donnons beaucoup de leçons de morale aux dirigeants hongrois ou polonais, nous menaçons maintenant les dirigeants italiens. À l'extérieur, nous sommes en froid avec nos amis marocains et nous avons des relations polaires avec beaucoup de pays africains. donc la suivante, madame la Première ministre : quelle initiative compte prendre votre gouvernement pour renouer le dialogue et essayer de trouver des solutions en Europe, afin de mettre en place des dispositifs efficaces ? La crise migratoire est une impasse qui nourrit

depuis plusieurs années, les questions migratoires sont au coeur de l'agenda européen. Malgré ses dangers, la Méditerranée centrale reste la voie la plus empruntée pour rejoindre l'Union européenne. Ces derniers jours, nous avons dû faire face à l'urgence après trois semaines, la situation à bord de l'devenait très préoccupante et appelait une prise en charge rapide. Dans ces circonstances, nous avons assumé pleinement notre devoir humanitaire. je vous le confirme, monsieur le sénateur, la France ne dévie pas d'une approche qui repose sur deux principes essentiels : l'humanité et la fermeté. Des mesures exceptionnelles ont été prises pour mettre en sécurité ces personnes, assurer le traitement le plus rapide possible des demandes d'asile et la reconduite de ceux qui ne relèvent pas de l'asile. Nous avons constaté que la solidarité européenne a été au rendez-vous, puisque onze pays européens ont accepté d'accueillir des migrants de l'et je voudrais devant vous, mesdames, messieurs Je veux saluer l'engagement de nos services publics, qui sont pleinement mobilisés pour apporter une réponse digne à ces situations humaines : le secrétariat général de la mer, la marine nationale, les préfets, l'Office Je veux enfin rendre hommage au travail de la Croix-Rouge française, qui a assumé les premières prises en charge. Notre responsabilité collective est de prévenir le renouvellement de telles situations. Ma conviction, c'est que la réponse ne saurait être seulement nationale, mais doit être aussi européenne. Européenne, d'abord, parce qu'un pays ne peut trouver seul les solutions à ces flux migratoires. Européenne, ensuite, parce que nous partageons un même espace, l'espace Schengen. Par conséquent, ce qui se passe à un endroit de cet espace nous concerne tous. Européenne, enfin, pour assurer le respect de deux principes cardinaux en la matière : la responsabilité et la solidarité. Cela suppose un cadre européen, avec des règles qui s'imposent à tous, et le respect des obligations internationales comme l'obligation du port sûr le plus proche. Force est de constater que l'Italie n'a respecté ni l'un ni l'autre. Concrètement, dans ce contexte, nous souhaitons agir dans trois directions principales. D'abord, la prévention des départs irréguliers en provenance d'Afrique du Nord. Cela passe par un renforcement des capacités maritimes des pays de départ et une plus grande efficacité collective en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière. Ensuite, la reprise des travaux sur les relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) impliquées dans le secours en mer en Méditerranée. Ces ONG sauvent des vies, accomplissent un travail important, mais une coopération plus fluide et plus transparente avec les pouvoirs publics est indispensable. Enfin, l'actualité confirme s'il en était besoin la nécessité d'avancer au plus vite sur la finalisation du pacte européen sur la migration Nous en avons fait une priorité lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et nous avons pu obtenir des avancées majeures. La présidence tchèque poursuit des discussions et nous souhaitons qu'un accord avec le Parlement européen puisse être rapidement trouvé sur ces sujets. En conclusion, nous sommes convaincus que ces enjeux requièrent une discussion politique. C'est pourquoi nous soutenons l'idée que soit rapidement convoqué à Bruxelles un conseil extraordinaire des ministres de l'intérieur afin d'examiner les réponses concrètes qui peuvent être rapidement apportées pour traiter le sujet dans toutes ses dimensions. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans quatre jours démarrera la coupe du monde de football, que nous pourrions appeler la coupe du monde de la honte. Jamais une coupe du monde n'aura suscité autant de malaises : corruption, désastres environnementaux, droits humains bafoués. sur le premier point, la justice finira bien par s'exprimer sur les conditions d'attribution. Au-delà de ces conditions, il s'agit d'une honte écologique. En plus de la climatisation des stades en plein désert, nous savons que ce ne sont pas moins de 160 vols quotidiens qui achemineront les supporters jusqu'à leurs hôtels. C'est une honte aussi pour les droits des femmes, des LGBTQI+, des minorités. Enfin, plus que d'une honte, il s'agit d'une catastrophe humaine. Les travaux pharaoniques ont mobilisé des milliers de travailleurs migrants. Exploités, ils ont bâti les stades dans des conditions insupportables : 6 500 d'entre eux y ont d'ailleurs laissé la vie. Alors que cet événement aurait dû être une fête populaire qui rassemble les peuples autour d'un sport, il se révèle un véritable désastre. Un tel scénario ne peut plus, ne doit plus se reproduire, que cela soit pour le football ou pour d'autres événements sportifs comme les jeux asiatiques d'hiver de 2029 qui auront lieu en Arabie Saoudite ... dans une région où l'on compte deux jours d'enneigement par an ministre, ne pensez-vous pas opportun que la France agisse pour la création d'une agence internationale chargée de contrôler l'attribution, mais également d'assurer le suivi des grands événements sportifs selon des critères de droits humains, sociaux et environnementaux ? La parole

croyons en la force de l'action diplomatique et la France oeuvre de manière continue par tous les canaux pour que, tant sur le sujet des droits humains que sur la question écologique, le Qatar non seulement consolide ses avancées qui sont d'ailleurs reconnues par l'Organisation internationale du travail

pour l'indemnisation des familles et des travailleurs. La Fifa a elle-même indiqué qu'elle s'associerait avec de nombreuses organisations internationales pour mettre en avant de grandes causes comme la lutte contre les discriminations, le développement durable, l'éducation, la santé. en suivi de mes demandes d'exemplarité, a pris elle-même des mesures pour s'assurer du respect des conditions de travail sur le camp de base de l'équipe de France. Ce n'est pas possible, ça ! Vous avez vu la lettre des Bleus qui ont souhaité rappeler leur attachement au respect de tous les droits humains et s'engagent à soutenir des ONG qui oeuvrent pour leur protection au travers de leurs fonds de dotation sénateur, vous avez raison : au-delà, ce Mondial doit nous amener collectivement à une plus grande responsabilité sociétale et à nous interroger sur le modèle des grands événements sportifs internationaux que nous souhaitons, ainsi que sur leur empreinte écologique. À cet égard, la Fifa est consciente de cette nécessité pour l'attribution des prochains Mondiaux de football. C'est ça ... À l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous montrerons aussi la voie. Vous le voyez, par-delà les polémiques, chacun s'engage dans la voie du nécessaire progrès.

Leur rôle, c'est de jouer au football. Que les supporters ne prennent pas d'acte politique, ce n'est pas grave ! Leur rôle, c'est d'encourager leur équipe. En revanche, que le Gouvernement ne prenne pas la mesure des choses, c'est plus regrettable ! Il n'est pas encore trop tard, madame la ministre. Nous pouvons marquer notre attachement aux droits humains et environnementaux par exemple par le port d'une tenue lors de l'entraînement d'avant-match, nous qui sommes, paraît-il, la nation des droits de l'homme. Très

et que le taux d'emploi atteint un niveau record depuis 1975, malgré les crises que nous traversons. Je vois bien que vous êtes tous favorables à ces éléments, mes chers collègues ! Ces résultats sont encourageants- et j'entends d'ailleurs vos encouragements ! -, même si les efforts doivent être intensifiés, notamment dans les secteurs en tension. en tension. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous le savons, c'est un enjeu majeur. Il est majeur d'abord, car il concerne 2,7 millions de bénéficiaires qui ont actuellement une reconnaissance administrative de leur handicap. Il est majeur ensuite, puisqu'il est foncièrement lié à notre volonté de bâtir une société plus inclusive, dans la continuité des engagements du Gouvernement et du Président de la République depuis 2017. Il est majeur enfin, car on ne peut pas accepter que le handicap soit un frein à l'accès à l'emploi de millions de concitoyens, mettant à mal leur émancipation et leur autonomie. Face à ce défi, le Gouvernement agit et les premiers résultats sont là. Le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap est à son plus bas niveau depuis cinq ans et le nombre d'apprentis a connu une progression de 175 % entre 2019 et 2021. Monsieur le ministre, le chemin est encore long. La 26 édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a débuté ce lundi, doit contribuer à changer le regard du handicap dans l'entreprise. Depuis 2018, le DuoDay ... En français, s'il vous plaît ! ... constitue un moment important pour faire tomber les préjugés et faciliter l'insertion des personnes Dans ce cadre, les 30 000 offres d'accueil sont autant d'occasions de créer de nouvelles opportunités professionnelles et de découvrir un environnement de travail. Monsieur le ministre, à l'occasion de ce rendez-vous incontournable pour démystifier le handicap dans l'entreprise, pourriez-vous nous indiquer les pistes que le Gouvernement envisage pour relever ce défi majeur en termes de cohésion sociale ?

hier sont une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque le taux de chômage, calculé au sens du Bureau international du travail (BIT), est passé de 7,4 % à 7,3 %, que cela vient corroborer la création de 84 000 emplois dans le secteur privé au cours du troisième trimestre et que le taux d'emploi des Français atteint 68,3 %, soit le meilleur niveau constaté depuis 1975. C'est rassurant, puisque, dans une période d'incertitude économique, l'économie continue à créer de l'emploi : de plus en plus de nos concitoyens retrouvent un emploi, qui plus est un emploi de meilleure qualité, puisque la part des contrats à durée indéterminée (CDI) a, pour la première fois depuis vingt-cinq ans, dépassé les 50 % de l'emploi total. C'est aussi une bonne nouvelle. Cette marche vers le plein emploi concerne tout le monde. Elle concerne bien évidemment aussi les travailleurs handicapés : le taux de chômage de ces publics est passé de 19 % à 13 % en cinq ans, mais il représente encore presque le double du taux de chômage moyen constaté. Nous devons donc continuer à agir.

les crédits consacrés aux entreprises adaptées passeront de 465 millions d'euros à 495 millions d'euros pour conforter le soutien de l'État aux entreprises adaptées. Nous reconduirons les expérimentations qui permettent la conclusion de contrats à durée déterminée dits CDD tremplin, qui permettent

permettant plus de fluidité et de passage vers l'économie ordinaire et reconnaissant plus de droits aux travailleurs dans les Ésat pour ainsi mieux les accompagner.

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le 25 novembre prochain, je veux souligner le caractère malheureusement massif des violences sexuelles et sexistes en France, comme le relève le rapport annuel 2022 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce, dans tous les secteurs- politique, médiatique, professionnel

Dans le domaine économique, les inégalités et discriminations subies par les femmes se renforcent encore : les femmes sont plus souvent confrontées à la précarité de l'emploi. on assiste à un recul des droits des femmes. Elles sont souvent les premières victimes de la répression des régimes dictatoriaux- on pense aux femmes afghanes -et c'est pour cela que les Iraniennes sont également les premières mobilisées contre le régime oppresseur. Aux États-Unis, depuis la décision de la Cour suprême remettant en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), les femmes sont en première ligne pour protester contre ce recul inacceptable de leur droit à disposer de leur corps. En France aussi, il y a un risque sur l'accès à l'IVG du fait de la désertification médicale et de la pénurie durable de gynécologues. Je regrette d'ailleurs que la majorité de droite du Sénat ait refusé l'inscription dans la Constitution du droit d'accès à l'IVG. Lorsqu'un droit fondamental des femmes est attaqué à l'échelle mondiale, on attend de la France qu'elle soit aux avant-postes pour le défendre ! Oui ! La question ! Le projet de budget pour 2023, marqué du sceau de l'injustice sociale et de la précarisation des classes populaires, ne parviendra pas à améliorer la situation. Madame la Première ministre, quand allez-vous dégager des moyens significatifs pour une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et résoudre enfin les difficultés quotidiennes vécues par nos concitoyennes ? La parole

et je suis fière d'appartenir à ce gouvernement, qui a permis de progresser comme jamais dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis 2017, quatre lois ont été votées pour mieux les protéger. C'est aussi +80 % de places d'hébergement d'urgence, 160 000 policiers et gendarmes formés, un déploiement massif des outils de protection des victimes- plus de 3 400 téléphones grave danger aujourd'hui

416 aujourd'hui, 600 prochainement - ; sans parler des 30 centres de prise en charge des auteurs pour prévenir la récidive. Grâce à la majorité parlementaire, les subventions au 3919 seront aussi augmentées- 5,9 millions d'euros en 2023, soit +400 soit +400 % depuis 2017. Le budget de mon ministère a doublé sous le précédent quinquennat et augmentera de 15 % l'an prochain.

pays de la Déclaration des droits de l'homme, doit être aussi celui des droits des femmes. Face aux montées des conservatismes, notre pays doit rester un phare pour les libertés de toutes les femmes. Vous pouvez compter sur ma détermination.

et prévoit que le Gouvernement adapte ces dispositions à l'outre-mer. Très tôt, les élus ultramarins ont pointé du doigt le niveau d'impréparation du gouvernement face à la mise en oeuvre de cette réforme outre-mer. C'est le cas pour Saint-Pierre et Miquelon où les acteurs sont plus que dans le flou. Certes, les

par mon cabinet, par mon ministère, mais également par la direction générale des outre-mer (DGOM) et la préfète sur place. Nous sommes évidemment très attentifs à la mise en place de ces dispositifs, car, vous le savez, à la suite d'un avis du Conseil d'État, la réglementation applicable en matière de formation professionnelle est celle du territoire national.

S'il apparaissait que certains points n'étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires ou, si certains devaient être encore précisés, les services de l'État proposeraient un accompagnement personnalisé pour finaliser ce dossier dans les plus brefs délais. pour objectif de favoriser l'agrément de l'association Opco 975 dès que cela sera possible. Vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, Akto met à disposition du territoire toute son expertise en matière d'ingénierie de formation et d'accompagnement des entreprises locales. Un accompagnement à la formation professionnelle est donc bien sûr assuré

reprise. Le contrat État-collectivité a été renouvelé à l'identique, avec des montants par conséquent maintenus. Monsieur le sénateur, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. La parole

J'ai pu observer dimanche, sur place, dans cette zone d'attente temporaire, ces entretiens, l'absence d'avocats, l'absence de traducteurs sur place, les bureaux ouverts aux quatre vents mettant à mal la confidentialité, l'absence de compréhension par le demandeur d'asile de ce qui se passait. Ce contexte dégradé ne permet pas d'émettre un avis. Les premiers entretiens de l'Ofpra ont débuté dimanche, ils sont aujourd'hui terminés. Hier, le ministre de l'intérieur a rappelé que le sort était fixé pour 148 personnes- 44 mineurs non accompagnés (MNA), 60 personnes acceptées, 44 refusées. Avez-vous des éléments sur la situation des 86 autres personnes rescapées ? Hier, le ministre de l'intérieur a fait des révélations troublantes. Au sujet des 44 personnes s'étant vu refuser le droit d'entrée au titre d'une demande d'asile, il a annoncé : « Elles seront évidemment reconduites. [ ...] J'ai pris contact dès hier avec mes homologues étrangers, à la demande de la Première ministre et du Président de la République. Quelle étrange chronologie annoncée par le ministre ! Vous le savez, les migrants qui se voient refuser l'entrée au titre de la demande d'asile doivent en recevoir notification et ont droit à un recours suspensif. Tant que tous ces délais ne sont pas expirés ou que le juge administratif n'a pas statué de manière définitive, ces migrants sont légalement toujours considérés comme demandeurs d'asile. Avant un refus définitif, tout contact avec leurs pays d'origine constitue une violation des conventions de Genève, un manquement grave au respect de la Convention européenne des droits de l'homme et, pis que tout, ils pourraient faire courir de nouveaux risques pour ces personnes. Madame la ministre, pouvez-vous justifier ces contacts précipités et contraires au droit avec ces pays ?

Comme vous le savez, le 11 novembre dernier, la France a pris la décision d'accueillir ce bateau qui naviguait en Méditerranée, avec à son bord 234 migrants secourus en mer

a rempli son devoir avec une triple exigence d'humanité, de sécurité et de fermeté. Concernant la situation de ces 234 migrants, je peux vous indiquer que, pour le moment, les démarches de l'Ofpra, tout comme les

Je vous confirme néanmoins que, à leur arrivée, toutes les mesures ont été prises afin d'apporter l'assistance sanitaire et médicale nécessaire aux passagers. Ceux-ci ont ensuite été placés dans une zone d'attente. Chacun d'entre eux fait l'objet d'un entretien individuel de sécurité avec les services spécialisés ainsi que d'un entretien administratif, comme vous l'avez rappelé, avec l'Ofpra. rappelé, avec l'Ofpra. Ceux qui peuvent obtenir l'asile seront accueillis partout en Europe, ce qui prouve bien, comme l'a dit la Première ministre il y a quelques instants, que la solution est européenne- et nous tenons à remercier nos partenaires de cette solidarité. La France a d'ailleurs demandé la tenue dans les tout prochains jours d'une réunion européenne à un niveau ministériel afin de traiter des suites de cette affaire. Madame la ministre, je n'ai pas eu de réponse à mes deux questions. Je le répète, accueillir dignement, c'est accueillir dans les règles et dans le respect des procédures. Accueillir dignement, ce n'est pas se réjouir et se féliciter d'avoir fait preuve d'humanité et, en même temps, publier des arrêtés préfectoraux interdisant les distributions de repas à Calais, après avoir été contraint de mettre en place des points d'eau. Accueillir, enfin, c'est secourir en Méditerranée, comme dans la Manche et comme dans les Alpes

La guerre en Ukraine et la remontée du prix des hydrocarbures ont achevé de convaincre ceux qui doutaient de la nécessité de poursuivre le développement de notre filière nucléaire française. L'Allemagne fait face à de graves difficultés pour n'avoir pas su diversifier suffisamment son mix énergétique. Elle paye aujourd'hui au prix fort sa dépendance au gaz russe et son abandon de l'atome. La France est dans une meilleure posture, même si elle doit faire face aux conséquences d'un certain nombre d'erreurs d'appréciation et d'anticipation. Plus personne ne doute à présent que le nucléaire soit l'une des principales composantes d'un mix énergétique souverain. Pour garantir à nos concitoyens et à nos entreprises une énergie fiable et abordable, il convient de moderniser notre parc. Veiller à la remise en état des réacteurs affectés par le phénomène de corrosion sous contrainte est une chose, mais la France doit aussi renforcer son parc existant en se dotant de nouveaux réacteurs. De nombreux territoires demandent à accueillir ces nouvelles installations. C'est le cas de la ville de Nogent-sur-Seine dans mon département de l'Aube, dont le site, initialement conçu pour quatre réacteurs, n'en accueille actuellement que Alors qu'un projet de loi sur le nucléaire est en préparation, nos territoires ont besoin de réponses quant au calendrier, aux critères d'éligibilité des sites et, plus généralement, madame la ministre, aux modalités de sélection des projets.

pour le pouvoir d'achat des Français, pour la compétitivité des entreprises, et nous le faisons évidemment pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans cette optique que nous avons conclu dès 2019 un contrat stratégique pour la filière nucléaire et engagé 0,5 milliard d'euros pour moderniser cette filière dans le cadre du plan de relance.

préciser notre mix énergétique. Vous aurez alors toutes les solutions sur la table. Le débat public sera lancé, et le délégué interministériel au nouveau nucléaire, qui vient d'être nommé, aura l'occasion de mettre en musique l'action des services de l'État pour soutenir le nouveau patron d'EDF dans ce projet industriel extraordinaire. C'est à ce moment-là que nous connaîtrons très exactement la trajectoire qui sera soumise à la représentation nationale. L'objectif est de recevoir nos premiers réacteurs en 2037.

À son bord, 230 migrants, dont une cinquantaine de mineurs, secourus en mer entre la Libye et l'Italie. Depuis des semaines, ce bateau naviguait sans destination. L'Italie refusait très fermement de l'accueillir, passant outre les conventions européennes. La France a dû se résoudre à l'accueillir. Pourtant, d'autres voies, alliant humanité et dignité, soutien et fermeté, étaient envisageables. Monsieur le ministre, vous annonciez vouloir réguler les flux migratoires. Vous annonciez aussi des négociations pour convaincre l'Italie d'accueillir le navire, alors qu'il était clair que son nouveau gouvernement refuserait. Finalement, vous avez ordonné son accueil et vous avez ouvert la voie aux passeurs. L'accueil de ce navire et la gestion de ces migrants créent un précédent d'une grande gravité. Du fait de votre manque de préparation et d'anticipation, des vices de procédure ont été soulevés. À cause du manque de moyens dont souffre la justice, leur situation n'a pas pu être examinée dans les temps. La conséquence est que, au moment où je vous parle, des migrants sont libres, sans que leur situation ait été examinée. Faute de moyens légaux de rétention, des mineurs ont déjà fugué. Votre incapacité à intervenir et, surtout, à anticiper les difficultés met gravement en cause la responsabilité du Gouvernement. Votre prédécesseur Gérard Collomb nous apprend qu'il a préféré démissionner plutôt que de se voir imposer par le Président de la République la création d'un grand centre d'accueil de migrants dans la ville de Toulon et de créer ce genre de situation et d'inquiétudes pour les habitants de Toulon et du Var. et du Var. Nous ne serons jamais insensibles, évidemment, à la souffrance des enfants, des femmes ou des hommes qui recherchent l'asile. Mais ne voyez-vous pas que, dans nos territoires déjà fragilisés et en manque de moyens, nous sommes aujourd'hui incapables de les assumer Nous ne voulons pas que nos côtes deviennent une nouvelle cible privilégiée pour les passeurs. Ma question est la suivante : monsieur le ministre, qu'allez-vous faire si de nouveaux bateaux se présentent ? À quoi les Toulonnais et les Français doivent-ils s'attendre ?

? Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, au fond, la réponse est assez simple. Il était de notre honneur d'accueillir ces migrants, et notamment les 44 enfants, qui se trouvaient en mer depuis quinze jours. Cela s'appelle tout simplement l'humanisme, une valeur dont la France s'honore depuis des siècles et qui fait son universalité.

Des décisions ont été rendues. Certaines font l'objet d'un appel. Vous le savez, la séparation des pouvoirs m'interdit de commenter ces décisions. Qu'allons-nous faire pour l'avenir ? Eh bien ! Nous allons nous

voyant les images de migrants massés à la frontière polonaise, a dit qu'il fallait les laisser crever de froid. Ce n'est pas l'option retenue par le Gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir.

La même année, à l'Assemblée générale des Nations unies, le Président de la République disait préférer une mobilité internationale choisie et non subie, au risque de faire monter les extrêmes. On connaît la suite de l'histoire : vendredi dernier, Emmanuel Macron donnait l'ordre d'accueillir les 230 migrants de l'à Toulon.

ont la plus grande difficulté pour se nourrir, se loger, se soigner, et en auront demain pour se chauffer- bref, pour survivre. En accueillant l', vous confondez humanitaire et appel d'air. En accueillant l', vous faites le jeu des passeurs. Sauver des vies en péril est une priorité, mais les bateaux de passeurs doivent être renvoyés dans les ports de départ Il est urgent que la France reprenne le contrôle de ses frontières. Il est urgent qu'il y ait une refonte de la politique d'immigration au niveau européen. Sinon, vous continuerez à dénaturer la France et à mettre les Français en danger. Oui, il existe un lien entre immigration et insécurité. Madame la ministre, combien faudra-t-il de Bataclan, de père Hamel, de massacres à Nice, de Lola, pour que vous preniez enfin

En quoi, monsieur le sénateur, êtes-vous fondé à faire le lien entre quelques dizaines de personnes en détresse en Méditerranée, dont une partie vient du Bangladesh, une cinquantaine sont des enfants mineurs, dont certains ont moins de 3 ans, et les attentats du Bataclan ? Qu'essayez-vous, monsieur le sénateur, d'instiller dans les esprits des Français ?

je ne crois pas que vous les regarderiez les bras croisés en disant qu'il n'y a pas de place sur notre territoire. Vous viendriez évidemment les aider ! Eh bien, la France peut s'enorgueillir de faire ce travail que chaque citoyen ferait à sa place, je l'affirme. La non-assistance à personne en danger n'est pas dans l'ADN de la France, de la République et du pays des Lumières, monsieur le sénateur

Monsieur le ministre de la santé et de la prévention, souvent tabous, les troubles psychiques concernent 13 millions de personnes : un Français sur cinq en souffre. Il s'agit du premier poste de dépense de l'assurance maladie, devant les cancers. La souffrance psychique conduit chaque année, en France, à 200 000 tentatives de suicide, avec 9 000 issues fatales, soit un taux de suicide parmi les plus élevés d'Europe. De nombreux décès sont évitables, Agnès Buzyn, ministre de la santé, reconnaissait « l'abandon de la psychiatrie ». Cinq ans après, rien n'a changé ! Monsieur le ministre, vous avez la responsabilité de la santé, mais aussi de la prévention. Un repérage précoce et une prise en charge adaptée amélioreraient la qualité de vie des patients. Vous me direz que, depuis 2022, l'assurance maladie rembourse les consultations de psychologue dès l'âge de 3 ans. C'est une avancée, mais elle est loin d'être à la hauteur des attentes. Parent pauvre de la médecine, aujourd'hui sinistrée, la psychiatrie publique manque d'argent et d'effectifs : 30 % des postes de psychiatres hospitaliers sont vacants et le nombre de postes d'infirmiers non pourvus a doublé entre 2019 et 2022. pour 2023 n'apporte aucune mesure pour sortir la psychiatrie de cette situation. Le nombre de patients augmente et augmentera en raison du covid-19. La prise en charge de L'usage des psychotropes et des mesures de contention augmente, dénoncé par les médecins eux-mêmes, qui n'ont pas d'autre choix. Les soignants sont en grande difficulté. Des enfants et leurs parents souffrent du manque d'accompagnement, alors que les files d'attente s'allongent dans les centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques. Depuis des années, les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Ils sont à bout. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie du Gouvernement pour répondre aux besoins de soins urgents en psychiatrie publique, notamment pour les enfants et adolescents ? Quel est votre projet de prévention sur le long terme pour les maladies psychiques ? La parole est à M. le ministre de la santé et de la prévention. Madame

(Ondam), en particulier pour l'hôpital, seront bénéfiques pour la psychiatrie. Sur le plan structurel, il y a plusieurs problèmes et deux combats à mener. Le premier combat se joue au niveau territorial, et consiste à travailler sur le maillage

Monsieur le ministre, depuis plusieurs semaines, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation vous a mis en garde contre des appels répétés de la mouvance islamiste visant à contourner la loi de 2004 qui, vous le savez, interdit les signes religieux à l'école. Cette mouvance encourage en particulier les jeunes filles, les réseaux sociaux, à porter des vêtements à connotation religieuse. Déjà, 720 signalements d'atteintes aux principes de laïcité dans les écoles ont été effectués par vos propres services. Depuis la rentrée scolaire, une vingtaine de jeunes filles portaient l'abaya au lycée Bourdelle de Montauban. La semaine dernière, nous avons appris qu'une enseignante de ce lycée a été placée sous protection policière après avoir fait une remontrance à l'une de ces élèves sur sa tenue. sa tenue. Cette élève a ensuite publié une vidéo de la scène, captée à l'insu de sa professeure. Monsieur le ministre, face à ces dérives répétées, à Montauban comme ailleurs, allez-vous clairement indiquer que le port de l'abaya est une atteinte délibérée au principe de laïcité et n'a pas sa place à l'école ?

portaient des abayas. La direction du lycée a engagé une procédure, qui commence par des échanges avec les élèves concernées et avec les familles,

Le proviseur ainsi que la professeure en question ont porté plainte. Une protection fonctionnelle a été accordée et la direction a travaillé en bonne intelligence avec la préfète

Monsieur le ministre, j'avais l'espoir que vous exprimiez une position un peu plus claire et ferme en réponse à ma question. Malheureusement, vous avez fait une réponse tout à fait ordinaire, et même administrative, ce que je n'attendais pas.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, il y a un an tout juste, j'interrogeais votre prédécesseur sur les leçons à tirer du tragique assassinat de Samuel Paty, dont nous célébrions il y a un mois le triste anniversaire. Ma question rejoint celle de mon collègue François Bonhomme, qui évoquait le département de Tarn-et-Garonne, mais le sujet est suffisamment important pour qu'on s'y attarde. vous en doutez bien, l'affaire du lycée Antoine Bourdelle de Montauban a très profondément choqué le corps enseignant. Monsieur le ministre, votre circulaire du 9 novembre dernier est supposée éclairer l'application de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. on constate tous les jours dans les établissements que cette circulaire laisse souvent enseignants et chefs d'établissement bien seuls face à des phénomènes de revendication religieuse et de radicalisation, en particulier face à de nouvelles manières d'affirmer son identité culturelle et religieuse, dont l'abaya est un parfait exemple. De quoi s'agit-il ? s'agit-il ? D'une longue robe, qui recouvre tout le corps sauf la tête et les mains. Bien que ce vêtement ne soit pas originellement de nature religieuse, ne soyons pas naïfs, son usage l'est clairement aujourd'hui. La loi de 2004 dispose que, à l'école, « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit Quelle est la doctrine de l'éducation nationale sur l'abaya au regard de la loi ? Vous n'avez pas répondu, monsieur le ministre. Ce vêtement est-il considéré comme une manifestation ostensible d'appartenance religieuse ? Malgré les précisions de la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté sur ce sujet, rien n'est clair. clair. L'incident de Montauban soulève une fois encore le problème de la formation et de la protection du corps enseignant, surtout au regard du danger représenté par les smartphones et les réseaux sociaux, véritables condensateurs de haine et de violence. Monsieur le ministre, la formation au métier d'enseignant comporte-t-elle des mises en situation concrètes, notamment pour les contractuels ? Leur apprend-on à réagir face à de telles provocations et agressions ? Sur la protection, a-t-on réellement avancé depuis l'assassinat de Samuel Paty ? La parole

Il faut avouer que, sur ce terrain-là, nos armes juridiques sont limitées. Je mets en garde les élèves contre ces influenceurs de mauvais aloi.

Parce que nous nous aventurerions sur un terrain extrêmement complexe. D'un point de vue juridique, l'abaya n'est pas simple à définir, et nous serions contournés la semaine suivante

question s'adresse à M. le ministre des armées. Nous avons bâti une partie de la dernière loi de programmation militaire sur le paradigme de la coopération européenne, et plus particulièrement franco-allemande. C'était effectivement une opportunité qu'il fallait saisir. Néanmoins, ce volontarisme dont la France a fait preuve se heurte aux dures réalités de la politique, de l'industrie et des intérêts. Depuis de longs mois, les signaux s'accumulent sur divers projets : l'avion de combat, le char, l'avion de patrouille maritime ... Les forces armées s'interrogent, comme d'ailleurs les industriels et comme les parlementaires, sur le calendrier, les conditions et, désormais, sur l'aboutissement même de ces différents projets. En ce qui concerne l'avion de combat, nous arrivons à une phase où chacun attend des garanties de l'État en matière de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre par Dassault Aviation, de prise en compte des besoins spécifiques de nos armées,

Premier fait : la France aura besoin d'un avion de combat du futur, parce que notre armée est une armée d'emploi, parce que nous entendons rester dans la course technologique et parce que ce système d'avion, mais aussi- je le rappelle -de combat, qui appartiendra aux forces aériennes et stratégiques, sera déterminant pour notre dissuasion. La France est engagée dans le Scaf, car elle y trouve son intérêt, avec ses partenaires allemands et- ne l'oublions pas -espagnols.

Les divergences entre les industriels se sont désormais largement estompées et, comme l'ont indiqué publiquement Éric Trappier et Guillaume Faury, l'accord entre les industriels est très proche.

L'objectif est que les contrats soient signés dès le mois de décembre prochain. Au-delà de la phase 1B, nous continuerons à préserver les intérêts stratégiques de la France, en ce qui concerne tant l'élaboration que l'exportation du Scaf. C'est important pour l'exportation, car en signant des accords de défense, c'est la parole de la France que nous engageons. Vous le savez, le ministre des armées est particulièrement attentif sur ce point. Je reprendrai, conclusion, ce qu'il a affirmé à de multiples reprises : il ne s'agit pas d'une affaire idéologique liée au couple franco-allemand. Il y aura, quoi qu'il en soit, un avion de chasse pour succéder au Rafale dans l'armée française.

-pour garantir leur supériorité dans les futures opérations et dans un monde où les avions de combat et les drones évoluent très vite, de même que les défenses antiaériennes. Pour la continuité de la

en France, des procédures d'exportation qui, me semble-t-il, sont robustes, suffisantes et efficaces. La parole est à M. Didier Marie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, dans un communiqué du 8 novembre dernier, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé que les producteurs d'énergie renouvelable allaient reverser 30,9 milliards d'euros au budget de l'État dans le cadre de la contribution au service public de l'électricité (CSPE). Cette contribution est exceptionnelle. C'est la première fois que l'État ne compense pas les charges de service public de l'énergie, mais au contraire, encaisse des recettes, exceptionnelles et inattendues, puisque les prévisions initiales envisageaient une dépense de 8 milliards d'euros pour l'État, soit un différentiel de près de 40 milliards d'euros. Cette inversion de tendance et les 30,9 milliards d'euros de recettes qui en découlent s'expliquent par l'augmentation des prix de gros de l'électricité par rapport aux tarifs garantis par l'État, dans le contexte énergétique et géopolitique que nous connaissons. À elle seule, la filière de l'éolien terrestre, parfois contraignante pour les communes et leurs habitants, apporte une contribution de 21,7 milliards d'euros. Comme l'indique la CRE dans sa communication, ces recettes supplémentaires devront financer le bouclier tarifaire. Alors que les élus locaux sont en première ligne face à l'explosion des prix de l'énergie, des matières premières et de l'inflation, comptez-vous utiliser concrètement cette manne financière pour soutenir les collectivités territoriales ? Bravo ! La parole

Accompagnez plus et mieux les collectivités dans leur projet de transition écologique. Cessez de vouloir contrôler les dépenses des collectivités ! Monsieur le ministre, il est inconcevable que, alors que vous enregistrez 30 milliards de recettes supplémentaires, de nombreuses communes soient contraintes de fermer des structures sportives et culturelles, de limiter l'éclairage public, d'augmenter les tarifs de restauration scolaire, de freiner leurs investissements. Monsieur le ministre, le compte n'y est pas ! Il est encore temps de corriger la copie. C'est ce que nous vous invitons à faire lors de l'examen du

comptes publics. Quand Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est présentée en mars 2020 aux élections municipales, elle avait proclamé deux engagements. Le premier était qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle. La France entière a alors constaté qu'elle n'avait pas tenu parole. Le second engagement a été fait la main sur le coeur : jamais elle n'augmenterait les impôts des Parisiens. Or non seulement elle n'a cessé de le faire depuis 2014, mais cette semaine, coup de grâce : les Parisiens ont appris d'une manière pour le moins cavalière qu'elle allait augmenter la taxe foncière de plus de 50 %, pour tenter de sortir Paris du chaos économique ! C'est encore La majorité de gauche avait pourtant hérité, ne vous en déplaise, d'une situation saine lors de l'alternance. Les Parisiens sont excédés. Les services publics ne sont pas à la hauteur d'une grande métropole européenne. Paris se déclasse Cela étant dit, il n'est pas envisageable, monsieur le ministre, que l'État en profite pour porter atteinte aux libertés communales. Il n'est donc pas sérieux de parler de mise sous tutelle. Cependant, il est temps que le Président de la République s'intéresse au coeur de la région capitale. Je souhaite donc que vous m'indiquiez, monsieur le ministre, par quelle mesure particulière le Gouvernement compte soulager les Parisiens, qui devront, de surcroît, faire des efforts dans la perspective des jeux Olympiques de 2024. est à M. le ministre délégué chargé des comptes publics. Madame la sénatrice Boulay-Espéronnier, quand je suis arrivé au ministère du budget il y a quelques mois, j'ai découvert que la Ville de Paris bénéficiait d'un arrangement avec la comptabilité publique, négocié à l'époque avec François Hollande, appelé système des loyers capitalisés.

Je vous raconte cela, madame la sénatrice, d'abord parce que j'ai décidé de mettre fin à ce système, qui était une véritable bombe à retardement pour les Parisiennes et pour les Parisiens, ensuite parce que cela dit tout de la gestion budgétaire de la Ville de Paris par Mme Hidalgo et son équipe. La réalité, c'est que Mme Hidalgo considère qu'elle est condamnée à taxer plus, parce qu'elle refuse de dépenser moins, de maîtriser ses dépenses et de mener des réformes. Marine Le Pen

l'État ne peut pas faire les réformes nécessaires à la Ville de Paris à la place de la Ville de Paris. La réalité, c'est que des réformes sont possibles et nécessaires. D'abord, appliquer strictement les 35 heures aux fonctionnaires de la Ville de Paris. Alors que la Ville a été condamnée à appliquer les 35 heures,

Tout cela pour vous dire, madame la sénatrice, que le Gouvernement et moi-même serons toujours aux côtés des Parisiennes et des Parisiens ... Il va falloir conclure ! ... ne serait-ce que pour conduire la Ville de Paris et lui indiquer les réformes nécessaires qui permettraient une gestion saine des finances publiques.

Les Républicains. Monsieur le ministre, il y a trois ans, le groupe Les Républicains marquait son profond désaccord avec la réforme du baccalauréat général et la disparition programmée de l'enseignement des mathématiques au lycée, voulue par Jean-Michel Blanquer. À l'époque, votre majorité refusait de voir le déclin du niveau global en mathématiques et le désintérêt dans notre pays pour cette matière. contraste était total avec la croissance quasi exponentielle des besoins technologiques dans notre pays pour répondre aux demandes de la société. Aujourd'hui, vous entreprenez un travail de déconstruction

Vous actez ainsi l'échec patent de la réforme susnommée et cela nous

Je me félicite, bien sûr, de ce retour à la raison un peu tardif, qui est de nature à consolider la culture scientifique du plus grand nombre. Mais la mise en oeuvre pratique est encore pour le moins confuse. Monsieur le ministre, disposerons-nous de suffisamment de professeurs pour assurer les cours à la rentrée ? Irez-vous au bout du raisonnement en permettant de choisir un troisième enseignement de spécialité en classe de terminale ?

partage bien entendu votre préoccupation et votre intérêt pour le niveau des mathématiques en France. Nous sommes dans une situation paradoxale : la France est un pays d'excellence en mathématiques- 13 médailles Fields -et, dans le même temps, il faut bien reconnaître que le niveau général de la population, notamment de la population scolaire, a baissé de manière importante dans cette matière ces dernières années. Tous les classements internationaux le démontrent. Nous avons donc réintroduit, en effet, une heure et demie de mathématiques dans le tronc commun

d'accrocher l'option maths complémentaires en terminale, aux côtés de la spécialité maths et des maths expertes. À cet ensemble, nous ajoutons un module

dans les filières scientifiques, particulièrement en mathématiques en classe de terminale. J'ai apporté des précisions en ce sens en disant que l'avenir de l'excellence mathématique en France reposait en grande partie sur les filles. Monsieur le ministre, trois ans : c'est le temps qu'il vous a fallu pour corriger votre copie et vos erreurs de calcul. Que de temps perdu avec cette politique du zigzag permanent qui caractérise finalement votre majorité depuis 2017 sur tant d'autres sujets ! Vous faites la démonstration, si j'ose dire, que la ligne du Gouvernement est en fait une spirale infernale dont les premières victimes sont nos jeunes générations, sacrifiées sur l'autel de vos atermoiements successifs. Il faut conclure ! Je ne me permettrai pas de vous commander, mais seulement de vous donner un conseil : la prochaine fois, n'hésitez pas à écouter la parole du Sénat.

prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion du mercredi 2 novembre 2022, un avis favorable, par 22 voix pour et aucune voix contre, à la nomination de M. Stanislas Bourron aux fonctions de directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis l'automne 2021, notre pays fait face à une inflation que nous n'avions pas connue depuis des décennies. À la faveur de la reprise de l'économie mondiale et en raison, depuis février 2022, de l'invasion de l'Ukraine, la vie chère met notre société à rude épreuve. Disons-le sans détour : la situation est particulièrement difficile et l'enlisement du conflit nous place dans une situation de grande incertitude- les missiles tombés hier sur le sol polonais nous l'ont encore rappelé. Oui, le contexte est sombre, mais notre choix est clair. Ce choix, c'est de lutter contre la vie chère pour protéger les Français et ce projet de loi de finances rectificative(PLFR) marque une nouvelle étape dans ce combat. C'est un combat que nous continuerons à mener l'année prochaine, car l'inflation devrait demeurer à un niveau élevé. Mais nous devrons le mener de façon différente, je veux bien sûr parler d'une approche plus ciblée dans les soutiens que nous apporterons, car l'équation des finances publiques d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle que nous connaissions durant cette parenthèse où l'argent- l'emprunt -semblait gratuit. Ce projet de loi de finances rectificative, qui n'est pas seulement un texte de fin de gestion, s'inscrit dans la continuité du paquet pouvoir d'achat que vous avez voté et enrichi cet été. Je vous le dis clairement : c'est une continuité que je revendique. Je la revendique, parce qu'elle constitue une réponse à l'urgence et nos compatriotes ne comprendraient pas qu'on les laisse démunis face aux prix qui augmentent. Je la revendique aussi, parce qu'elle a produit des résultats : la France est le pays de la zone euro où l'inflation est la plus contenue. Avant de vous présenter les grandes lignes de ce texte, il me semble utile de vous dire un mot sur la situation de l'économie française en cette fin d'année 2022. Vous le savez, les prévisions adossées à ce deuxième projet de loi de finances rectificative font état d'une croissance de 2,7 % cette année, un chiffre jugé crédible par le Haut Conseil des finances publiques. Pour ma part, au-delà des prévisions, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si nous mettons tout en oeuvre pour atteindre notre objectif. Il est évidemment trop tôt pour dire avec une absolue certitude si nous y parviendrons, mais ce qui me semble incontestable, c'est que le texte que nous vous présentons aujourd'hui intensifie notre combat contre la vie chère et qu'il permettra donc à l'économie française de mieux tenir le choc.

publiques, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre économie résiste admirablement en cette fin d'année 2022. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien ou de verser dans l'autosatisfaction, mais simplement de savoir distinguer les signes encourageants malgré l'incertitude. La réalité, c'est que nous sommes au coeur de la tempête, mais que cette tempête ne nous emportera pas. Non, elle ne nous emportera pas, car nous pouvons compter sur des fondamentaux solides. Je souhaite à cet égard rendre hommage

notre pays, qui tiennent bon malgré les aléas, les difficultés et la hausse des factures, à ces entrepreneurs qui continuent d'investir, d'inventer, d'embaucher. Bref, ce que je veux saluer, c'est cette France qui résiste et qui ne cède pas un pouce de terrain à la morosité.

L'investissement des entreprises a crû de 2,3 % ce trimestre, tandis que la consommation des ménages s'est maintenue. La situation de l'emploi constitue un autre indicateur positif, puisque les créations d'emplois sont restées dynamiques au troisième trimestre. Encore au mois de septembre, nous avons comptabilisé 60 000 chômeurs de moins. S'agissant de ce qui nous attend pour ce quatrième trimestre, les signaux et indicateurs dont nous disposons sont plutôt favorables, qu'il s'agisse de l'activité, des intentions d'embauches ou de l'investissement des entreprises. Bien entendu, le niveau élevé d'inflation suscite des inquiétudes du côté des ménages comme des chefs d'entreprise. La hausse des prix a en effet rebondi à 6,2 % en octobre après 5,6 % en septembre. Pour autant, ce niveau reste cohérent avec la prévision adossée à ce deuxième PLFR, c'est-à-dire une inflation de 5,3 % en moyenne annuelle, jugée elle aussi crédible par le Haut Conseil des finances publiques. Ne nous voilons pas la face : nous avons l'inflation la moins élevée de toute la zone euro, mais la dynamique de hausse des prix fait encore des dégâts. Le texte que nous vous présentons aujourd'hui permet d'assurer le financement de mesures qui vont changer le quotidien des Français, tout en procédant à un certain nombre d'ajustements dans une logique très classique de fin de gestion. Comme le PLFR de juillet, ce texte traduit d'abord une volonté de soutenir et de protéger. Pour ma part, il me semble qu'une large majorité peut se retrouver dans cet objectif. D'ailleurs, ce texte a été adopté

Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est une rallonge de 2,5 milliards d'euros. Un petit mot sur la dette ? Cette rallonge va notamment permettre d'aider 12 millions de ménages à payer leurs factures énergétiques, qu'ils se chauffent au gaz, à l'électricité, au bois ou au fioul. Avec ce texte, nous mettons 1,8 milliard d'euros sur la table pour financer le chèque énergie exceptionnel. Concrètement, c'est un versement de 100 euros ou de 200 euros qui sera effectué d'ici la fin de l'année. J'en profite pour rappeler que la première loi de finances rectificative a prévu un budget de 230 millions d'euros pour aider les ménages qui se chauffent au fioul. Cette aide commence à être versée, elle se traduit par l'attribution d'un chèque de 200 euros pour les ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie et de 100 euros pour les ménages des troisième Il y avait un angle mort : les ménages qui se chauffent au bois. Il fallait corriger cela, car ils sont quand même 3,4 millions dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale pour mettre en place une aide exceptionnelle pour les ménages qui utilisent le bois comme mode de chauffage. Au-delà des 230 millions que nous avons ainsi débloqués pour alléger la facture d'une partie de nos compatriotes, nous voulons également- je le dis avec fermeté -lutter contre l'opacité du marché du bois de chauffage et les comportements spéculatifs qui nuisent à des ménages qui sont déjà parfois en grande difficulté. Ce texte finance un autre choix que nous avons fait depuis le 1 avril : celui de soutenir les automobilistes. Vous le savez, la Première ministre avait annoncé une prolongation jusqu'à la mi-novembre de la ristourne de 30 centimes par litre pour tenir compte du blocage des raffineries et des difficultés d'approvisionnement dont ont pâti nos compatriotes.

Vous le voyez, ce PLFR est un texte dont les mesures contribueront à améliorer le quotidien de nos compatriotes dans ces moments difficiles. C'est aussi un texte de soutien aux opérateurs de l'État face à l'envolée des prix de l'énergie- je pense notamment aux universités, aux établissements de recherche et aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous). Nous avons prévu une enveloppe de 275 millions d'euros, immédiatement débloquée au bénéfice des opérateurs du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

nos soldats. Ainsi, 2,5 milliards d'euros sont mis sur la table pour aider les Français et certains opérateurs de l'État à faire face au choc énergétique. Mais, avec ce texte, il ne s'agit pas seulement de parer à l'urgence, il s'agit aussi de procéder à un certain nombre d'ajustements de fin de gestion avec le souci permanent de tenir les comptes publics. globale, les ouvertures de crédits auxquelles nous procédons pour assurer de nouvelles dépenses, de l'ordre de 5 milliards d'euros, sont compensées par des annulations de crédits d'un montant identique.

La principale de ces ouvertures de crédit, à hauteur de 2 milliards d'euros, permet de poursuivre le développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce sont ainsi 2 milliards d'euros de crédits que nous ouvrons pour financer France compétences ... Ce n'est pas la première fois ! ... afin d'aider chaque Français à construire son avenir professionnel. Ces 2 milliards d'euros sont la traduction du formidable défi que nous sommes en train de relever sur l'apprentissage après des années où nous avions fini par croire que cela était impossible.

Autre ouverture significative de crédits : 1,1 milliard d'euros pour la mission « Défense » afin de financer le soutien militaire que nous apportons à l'Ukraine. Dernière ouverture de crédits que je souhaite mentionner dans ce propos liminaire : celle de 450 millions d'euros pour prolonger le financement des mesures d'indemnisation des crises agricoles survenues cette année.

En contrepartie, nous procédons à des annulations de crédits d'un montant équivalent qui ont pour effet de couvrir intégralement les ouvertures que je viens de présenter. J'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir durant ce débat. Je vous disais que notre premier objectif est d'aider l'économie française à absorber le choc.

Je le disais, hors dépenses exceptionnelles liées à la crise de l'énergie, nous vous présentons aujourd'hui un texte sans ouverture nette de crédits. Notre pays, malgré les aléas, ne cède pas un pouce de terrain au laisser-aller budgétaire.

mesdames, messieurs les sénateurs, cette rallonge anti-inflation, nous la finançons tout en poursuivant notre objectif de maîtrise des comptes publics. Ainsi, 2022 n'est pas seulement l'année du combat contre la vie chère, c'est aussi l'année du combat pour des comptes bien tenus. Cette maîtrise des comptes est possible grâce à une économie qui résiste et à l'engagement et au travail de chacun. Avec ce projet de loi de finances rectificative, nous aidons les Français à se chauffer et à se déplacer, nous aidons nos étudiants et nos chercheurs à travailler dans de bonnes conditions, nous poursuivons le financement de la bataille en faveur du plein emploi et nous assumons notre choix de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien. Ces objectifs, je pense qu'une immense majorité des Français les soutient et, parce que les Français n'ont tout simplement pas les moyens d'attendre, il nous revient d'agir au service de l'intérêt de notre pays. La parole

que l'on qualifie généralement de PLFR de fin de gestion. Le principal objectif de ce texte est de procéder à divers ajustements, ouvertures et annulations de crédits sur le budget de l'État. J'y reviendrai, mais en réalité l'examen à l'Assemblée nationale a conduit à aller plus loin, monsieur le ministre, en introduisant aussi cette année des mesures fiscales pérennes, revenant sur une pratique établie depuis 2018.

La prévision retenue par le Gouvernement se situe dans la borne haute du consensus des économistes, mais elle ne paraît pas pour autant inatteignable. Le ralentissement de l'activité au troisième trimestre plaide plutôt pour une croissance plus proche de 2,5 %.

Cette légère amélioration, qui laisse tout de même nos comptes publics dans un état plus que préoccupant, s'explique à la fois par des anticipations de recettes plus plus importantes en matière de prélèvements sociaux et d'impôt sur le revenu et par des dépenses moindres liées à des économies de constatation. Avec un peu plus de 172 milliards d'euros, le déficit budgétaire de l'État serait finalement supérieur

millions d'euros, principalement par une augmentation des dépenses du budget général. Dans les grandes masses, l'amélioration de la prévision de déficit par rapport à la loi de finances rectificative s'explique d'abord par la révision à la hausse des recettes nettes et du moindre niveau attendu du prélèvement sur recettes à destination de l'Union européenne. Mais l'amélioration du solde provient également d'une consommation moindre de crédits reportés, puisque seuls

sur le programme 134, « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie », mais ce programme dispose toujours de 4,5 milliards d'euros non consommés, car de très importants crédits ont été ouverts en cours d'année pour financer les dispositifs d'aide aux entreprises face à l'inflation et ont été très peu utilisés. Ces crédits vont probablement être massivement reportés sur 2023. l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, comme la Cour des comptes, monsieur le ministre, cette pratique n'est pas satisfaisante : les reports massifs de ce type ne devraient plus être pratiqués.

Quoi qu'il en soit, le déficit demeure considérable, puisqu'il serait à peu près identique aux niveaux atteints en 2020 et 2021, soit deux fois plus que celui constaté au cours des années 2011 à 2019. Le projet de loi de finances rectificative suppose toutefois un niveau exceptionnel de dépenses en fin d'année avec une dégradation de près de 25 milliards d'euros dans les trois derniers mois de l'année. Il est vrai que des dépenses importantes sont prévues au titre, notamment, des mesures de protection contre l'inflation, mais il est bien possible que, une nouvelle fois, des crédits importants demeurent non utilisés à la fin de l'année. En tout état de cause-

Le niveau des recettes ne varie pas de manière fondamentale malgré de bonnes nouvelles qui se poursuivent sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Mais comme je l'indiquais à l'instant, ce collectif budgétaire contient aussi cinq articles comprenant des dispositions fiscales dont la portée va au-delà de l'exercice 2022.

La commission des finances propose toutefois de supprimer l'article 9 C relatif à la répartition entre les collectivités territoriales et leurs groupements du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les

Pour les années à venir, comme nous l'avons prévu en révisant la loi organique relative aux lois de finances, il conviendra de revenir à une séparation nette entre le collectif budgétaire qui ajuste les crédits en fin d'année et le projet de loi de finances qui prépare le budget et les dispositions fiscales Mais c'est bien du côté des dépenses que ce PLFR apporte le plus de modifications avec des ouvertures qui dépassent de loin les annulations.

Pour autant, l'équilibre financier pérenne de cet opérateur n'est toujours pas assuré. Monsieur le ministre, une trajectoire soutenable pour le financement de la formation professionnelle Le niveau élevé de l'inflation et plus particulièrement des prix de l'énergie reste l'une des principales causes d'ouvertures de crédits. Il s'agit par exemple du chèque énergie exceptionnel, mais aussi de la prolongation de la remise carburant que vous avez évoquée, monsieur le ministre.

Un nouveau programme, doté de 1,4 milliard d'euros, doit compenser à la sécurité sociale le coût des dons de vaccins à des pays tiers et aussi lui reverser une partie des sommes reçues de l'Union européenne dans le cadre du plan de relance au titre du volet investissement

S'agissant, enfin, des effectifs, la régularisation opérée par le texte conduit à une hausse de 1081 emplois. Je ne vous cache pas que la commission des finances s'en est étonnée, notamment s'agissant des 53 emplois créés au sein des services de la Première ministre, y compris pour le Conseil national de la refondation, même si le nombre reste symbolique. En conclusion, la commission des finances propose d'adopter les mesures proposées par le Gouvernement

plus favorable, de MaPrimeRénov'. Nous proposerons également l'ouverture de deux enveloppes destinées à renforcer les moyens alloués, d'une part, à la réfection des ponts, notamment des petites communes, avec 60 millions d'euros supplémentaires,

Je ne sais pas si vous avez emprunté l'hélicoptère bleu ou l'hélicoptère rouge, comme dans la célèbre émission télévisée, mais vous avez remporté la chasse au trésor.

Comme je l'ai souligné en commission des finances, à tout prendre, je préfère qu'il y ait des trésors cachés plutôt que des déficits cachés. Vous avez gagné cette chasse au trésor et nous arrivons à équilibrer ce second PLFR sans faire appel à l'emprunt, ce qui est rare, et en offrant un soutien aux entreprises et aux particuliers qui sont frappés de plein fouet par la crise énergétique.

le contexte géopolitique nous invite à rester prudents sur les prévisions de croissance économique, soit +2,7 % du PIB pour 2022, légèrement plus optimistes que lors de la première loi de finances rectificative, mais inférieures aux +4 % prévus en 2021. Le Haut Conseil des finances publiques estime que les prévisions de croissance et d'inflation du Gouvernement restent crédibles- « un peu élevées » sans être « hors d'atteinte » -, les niveaux d'inflation et de déficit étant quelque peu sous-estimés.

L'article 3 traduit l'incidence sur l'équilibre budgétaire en 2022 des dispositions du présent PLFR et de la réévaluation des recettes. Le solde budgétaire s'améliore légèrement

L'article 6 prévoit 439 millions d'euros en autorisations d'engagement et 442 millions d'euros en crédits de paiement, principalement pour les avances aux collectivités territoriales. Quant à l'article 7, il prévoit prévoit 907 équivalents temps plein d'autorisations d'emplois de l'État pour renforcer les dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales et la justice de proximité.

un chèque énergie exceptionnel, bien peu exceptionnel, tant cette année d'élection présidentielle aura été l'année des chèques. Ainsi, 12 millions de foyers, sur le critère du revenu fiscal, seraient concernés.

Certes, la recherche d'équité est difficile, mais on touche là aux limites de l'exercice du chèque. On peut en dire autant de la prolongation de la remise sur le carburant pour deux semaines Inquiétante également est la rallonge de 2 milliards d'euros consentie à France compétences. Elle survient en effet après une première rallonge du même montant dans le premier PLFR et précède un effort d'encore 2 milliards d'euros annoncé dans le PLF 2023, qui s'ajoute aux 3,5 milliards d'euros en supplément pour l'augmentation des contrats d'apprentissage.

Sachant qu'un tiers des dépenses de cet organisme est relatif à la formation, et considérant le catalogue parfois surprenant de ces formations, je crois qu'il y a là matière à contrôle parlementaire. Les autres dépenses sont plus légitimes : activité opérationnelle des forces armées, aides aux agriculteurs, équipements militaires de l'Ukraine, pour un total global de 7,5 milliards d'euros de dépenses nouvelles. En regard, En regard, il y aurait 5 milliards d'euros d'annulations de crédits, notamment 2 milliards d'euros au titre des PGE et 500 millions d'euros au titre des dépenses accidentelles, dont nous avions dit qu'elles étaient surestimées. Voilà pour le texte, mais c'est le contexte qui me paraît le plus intéressant. Nous devrions terminer l'année 2022, certes en amélioration par rapport à l'estimation initiale,

% du PIB, nous avons le niveau de prélèvements obligatoires le plus élevé des 38 pays de l'OCDE -en compagnie de la Finlande et du Danemark, il est vrai. Cela porte à relativiser le discours triomphaliste du Gouvernement en la matière. Comment peut-on parvenir à un tel déficit quand on a un taux si élevé de prélèvements obligatoires ? En laissant filer les dépenses publiques, bien sûr ! Celles-ci augmentent, même diminuées des dépenses exceptionnelles. Le taux de dépense publique en France, en 2022, demeure plus important qu'en 2012, 2017 et 2019. Il est surtout le plus élevé de l'Union européenne. européenne. des administrations de l'État, les collectivités territoriales ont pour leur part, et comme toujours, joué le jeu de la maîtrise de la dépense publique, puisque, en 2022, le déficit des administrations publiques locales est égal à zéro

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénat a exigé que l'État fasse autant d'efforts que ceux qu'il demande aux collectivités, en alignant les deux trajectoires budgétaires dans la loi de programmation des finances publiques. Le Le fonctionnement courant de notre État est donc financé par la dette de la France, l'une des plus élevées de l'Union européenne. En 2012, à la fin du quinquennat Sarkozy, notre pays avait un endettement de 90,6 % du PIB, exactement dans la moyenne de la zone euro, qui était de 90,7 %. En 2022, à la fin de cette année, après les quinquennats Hollande et Macron, la France a un endettement de 111,5 % du PIB, contre 95 % dans la zone euro. L'Allemagne, quant à elle, est à 66 Si, en face de ces records, très négatifs, bien évidemment, en matière de dette, de dépenses publiques, de prélèvements obligatoires, nous constations un faible taux de chômage, une vraie réindustrialisation, avec une balance de commerce extérieur favorable grâce à l'investissement, des services publics de bon niveau concourant au bien-être quotidien des Français, peut-être verrions-nous ces chiffres d'un autre oeil. Mais, là aussi, le diagnostic est sombre.

Et encore cette baisse est-elle en partie due à la mise en formation de nombreux demandeurs d'emploi. que des centaines de milliers de postes sont vacants dans de très nombreux secteurs, y compris dans l'emploi public, nous comptons quasiment 3 millions de chômeurs de catégorie A. Enfin, le déficit commercial bat tous les records et dépassera probablement 200 milliards d'euros au 31 décembre 2022. Il avait déjà atteint plus de 143 milliards d'euros

Quant aux services publics, leur état est peut-être encore plus préoccupant que les chiffres calamiteux des indicateurs des finances publiques. Si l'on hésite sur le sort de l'hôpital, c'est qu'on ne sait pas trop dire s'il a déjà craqué ou s'il va craquer

Les ministères et leurs administrations sont tellement efficaces qu'il a fallu, en 2021, recourir à des cabinets de conseil pour éclairer les choix stratégiques, pour un montant supérieur à 1 milliard d'euros.

Pourtant, ce PLFR, dans son article 7, augmente le plafond d'emplois : plus de 900 équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) pour l'État, plus de 170 pour ses opérateurs. Plus de fonctionnaires, une masse salariale qui augmente en 2022 et toujours moins de services dans nos territoires

Ce bilan aurait dû sonner comme une alarme pour le Gouvernement, mais il n'en est rien. Mes chers collègues, quand nous regardons la situation, nous nous désolons, et quand nous nous comparons avec nos voisins, la désolation est encore plus complète, à la lumière des quelques chiffres que je viens d'exposer.

Certes, ce texte remplit sa mission de collectif budgétaire de fin de gestion, mais il contient également plusieurs mesures nouvelles. Les principales sont dictées par l'urgence de la situation que nous vivons et concernent l'inflation. à atténuer les coûts liés à la hausse des prix de l'énergie. C'est notamment le cas du chèque énergie exceptionnel, d'un montant de 100 ou 200 euros, qui sera versé aux ménages les plus modestes. Ce dispositif est bienvenu, car il permet de mieux cibler les efforts budgétaires sur ceux qui en ont le plus besoin en complétant les dispositifs mis en place antérieurement. Force est de constater que l'inflation ne frappe pas tous les Français avec la même intensité. Elle pénalise les ruraux plus que les urbains,

Il importait également que ce dispositif concerne bien toutes les sources d'énergie. C'est pourquoi la création d'une aide de 230 millions d'euros pour les ménages se chauffant au bois, avec des calquée sur le chèque exceptionnel fioul, est une avancée que je soutiens pleinement. En complément, j'ai proposé un amendement pour étendre le bénéfice du taux de TVA réduit aux pellets, aux granulés bois et aux plaquettes. Le prolongement de la ristourne sur le carburant à la pompe permet aussi de répondre aux préoccupations des Français qui subissent de plein fouet la hausse des prix. En effet, même si ce dispositif n'est pas ciblé, puisqu'il n'est pas soumis à des conditions de ressources, il vise avant tout ceux de nos compatriotes qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture. Cette mesure évite la complexité d'un accès sous conditions et s'adresse prioritairement à la ruralité. C'est un facteur de cohésion sociale en ces temps de forte inflation. Néanmoins, nous avons déjà pu constater plusieurs formes de détournement de cette mesure. C'est particulièrement le cas dans le Grand Est, où nous voyons de nombreux transfrontaliers, Belges, Luxembourgeois, Allemands ou Suisses venir en France pour bénéficier des prix réduits grâce aux impôts des Français. Nous devons y remédier en ciblant mieux ces aides.

Il importe que nos dispositifs ciblent davantage les travailleurs. Dans notre département de la Meuse, cher Gérard Longuet, ... Eh oui ! ... 82 % d'entre eux prennent leur voiture pour aller travailler. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Nous devons rassurer les Français sur notre volonté de mieux valoriser le travail. J'y insiste, la flambée des prix de l'énergie fragilise nos concitoyens qui doivent prendre chaque jour leur voiture pour se rendre à leur travail, en particulier dans les territoires ruraux. Ce PLFR a aussi été enrichi de plusieurs propositions de l'Assemblée nationale. Nombre d'entre elles nous semblent pertinentes, comme les ajustements apportés au dispositif MaPrimeRénov', ou encore l'extension de l'exonération permanente de taxe foncière pour les bâtiments ruraux affectés à un usage agricole. Je pense également à la réforme de l'Ifer pour le photovoltaïque au bénéfice des communes. Cette mesure reprend une proposition que notre groupe défendait depuis plusieurs années. Certes, elle n'a sans doute pas sa place

Notre groupe salue l'augmentation des effectifs du ministère de la justice, ... Le nôtre aussi ! ... en espérant que cela améliore l'efficacité et la célérité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire national. C'est une forte et légitime attente de nos concitoyens. Néanmoins, d'autres augmentations interrogent. Toutes ne répondent pas à une urgence, et devraient plutôt être être intégrées au PLF. Au-delà de ces réserves, et pour l'essentiel des dispositions, nous considérons que ce texte va dans le bon sens et permettra de renforcer le pouvoir d'achat des Français.

Je souligne plus précisément les 275 millions d'euros pour aider les universités et les opérateurs de recherche à payer leurs factures énergétiques. Il contient aussi un nouveau chèque énergie bienvenu, qui cible les ménages les plus modestes, et des avancées que l'on doit au travail parlementaire, preuve de son utilité : 230 millions d'euros d'aides pour les ménages qui utilisent du bois domestique comme source de chauffage, le soutien à la filiale presse

Les boucliers tarifaires sont utiles pour panser les plaies face aux multiples crises que nous traversons, mais ils sont inefficaces, coûteux et même inéquitables face à la bifurcation écologique, urgente et nécessaire.

en SUV ? Et pourquoi faire porter cet effort uniquement par le budget de l'État, quand les pétroliers dégagent des profits indécents ? Pis encore, cette mesure d'urgence va à l'encontre d'une autre urgence, vitale celle-là : réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

cher collègue ... Ciblez, monsieur le ministre, aidez ceux qui n'ont pas le choix et appelez la contribution de ceux qui accumulent dividendes et biens. Comme seconde illustration, je prendrai la situation dans laquelle sont placés les élus locaux.

La DGF n'est pas une subvention, mais une dotation pour services rendus. Indexez-la sur l'inflation, renoncez à la suppression de la CVAE et imposez un tarif réglementé de l'énergie pour toutes les collectivités. Je présenterai des amendements en ce sens. Les élus des collectivités sont assez intelligents pour prévoir et décider en responsabilité. Il faut toutefois leur donner la possibilité

en sorte que chaque décision ponctuelle porte en elle les choix de la résilience durable. À l'issue de la COP27, le Président de la République sera une fois encore dos au mur. Il doit agir concrètement et fortement pour la transition écologique et sociale. Le saupoudrage, les mesures ponctuelles ne suffisent plus. Il faut accélérer pour organiser la résilience de notre pays. Ce PLFR, hélas, ne procède toujours pas de cette logique.

tenir compte des crises survenues pendant l'année, les crédits sont ajustés en fin d'exercice, avec des ouvertures compensées à hauteur de 5,4 milliards d'euros : +2 milliards d'euros pour France compétences ; +500 millions d'euros pour le pour le ministère du travail au titre de l'actualisation de la prévision sur les compensations d'exonération de cotisations sociales ; +1,1 milliard d'euros pour les forces armées françaises en raison des surcoûts opérationnels, dans le contexte de guerre que nous connaissons. Sans oublier les 450 millions d'euros prévus au titre des mesures d'indemnisation économiques liées à la conjoncture ou encore les 200 millions d'euros ouverts sur le programme du ministère de la santé et de la prévention permettant de financer l'indemnité exceptionnelle versée aux salariés, autoentrepreneurs et indépendants. Ce sont autant d'ajustements de crédits nécessaires et bienvenus face à l'ampleur de l'inflation et aux conséquences de la crise énergétique. Néanmoins, mes chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative, d'apparence traditionnelle,

Ce second PLFR finance également la prolongation de la remise sur le carburant, à hauteur de 460 millions d'euros. Certes, depuis hier, la remise à la pompe n'est plus que de 10 centimes, mais je tiens à rappeler deux choses

». Ce texte est également inédit par les conditions de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, dans le contexte politique que nous connaissons tous. Force est de constater que des amendements provenant des multiples bancs de l'opposition ont été adoptés. C'est ainsi que 8 millions d'euros viendront aider les communes qui versent des primes aux soignants des centres municipaux de santé, ou que 40 millions d'euros de crédits supplémentaires aideront les associations d'aide alimentaire à faire face face à l'augmentation du nombre de leurs bénéficiaires. Finalement, ce PLFR démontre que, lorsqu'un dialogue apaisé et constructif s'installe, le Parlement peut travailler sereinement sur un texte budgétaire et l'adopter, même en l'absence de majorité absolue. Nos collègues députés ont débattu dans un état d'esprit constructif. J'espère, mes chers collègues, que notre assemblée en fera tout autant, si ce n'est davantage

objectif est de prévenir les effets de seuil que nous connaissons tous dans nos communes, en permettant, pour celles d'entre elles dont la baisse d'épargne brute est comprise entre 20 % et 25 %, la compensation d'une fraction réduite des dépenses d'approvisionnement.

Ce texte n'est qu'un exercice de fin de gestion permettant d'actualiser nos prévisions macroéconomiques, de corriger les ouvertures de crédits et de prendre des mesures d'urgence à effet immédiat. Il se contente donc, pour sa majeure partie, de prolonger ou d'adapter des dispositifs d'aide existants, le temps de terminer l'exercice 2022. Avant de détailler les points de divergences qui éloignent notre groupe de ce collectif budgétaire de fin d'exercice, je tiens néanmoins à dire que certaines aides prévues dans le texte vont dans le bon sens. Je pense notamment aux aides accordées aux universités pour payer leur facture énergétique, aux armées pour le carburant, ou aux agriculteurs pour faire face aux conséquences des diverses crises qu'ils subissent.

Dans un contexte international porteur de guerre, au lendemain d'un événement, en Pologne, dont on ne sait rien, mais dont on imagine tout, il semble nécessaire de maintenir un rapport de force suffisant, avec toujours pour seul objectif la recherche de la paix. Mais revenons à la France, car quelques chiffres devraient nous interpeller : un Français sur dix dépend de l'aide alimentaire ! Dans le même temps, une personne sur cinq a froid dans son logement et 12 millions de nos compatriotes subissent la précarité énergétique.

et ils ne cachent que trop mal votre absence de vision quant au nécessaire déploiement d'une politique visant à recouvrer notre souveraineté énergétique et à effectuer la bifurcation écologique tant vantée durant la COP27 en Égypte.

Depuis 2020, le Président de la République utilise cet argument pour mieux justifier son inaction en la matière, mais le temps presse : nous comptabilisons plus de 7 millions de passoires énergétiques en France. Je rappelle que les rénovations énergétiques ont deux vertus

souligner le renforcement des crédits alloués aux associations oeuvrant à l'aide alimentaire. Grâce au travail de mes homologues socialistes à l'Assemblée nationale, 40 millions d'euros supplémentaires seront débloqués afin de permettre à ces

Nous sommes bien conscients que tout cela a un coût que nous n'ignorons pas. Nous pensons même que ce coût doit être supporté par tous, parmi lesquels je compte bien évidemment les profiteurs de crises qui réalisent des superprofits. Ces profits sont, en grande partie, le produit de rentes ; ils ne découlent nullement d'un quelconque génie entrepreneurial si souvent vanté pour légitimer les salaires astronomiques de certains dirigeants. Nous considérons que cette contribution doit permettre une juste répartition de la richesse dans ce pays et nous veillerons, dans le débat sur le budget pour 2023, à ce que cette mesure d'équité économique trouve une issue favorable. Enfin, je note une nouvelle fois, monsieur le ministre, que vous semblez découvrir en fin d'exercice près de 5 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. J'entends votre volonté, que nous pourrions presque louer, de ne pas faire de projections de recettes trop favorables en début d'exercice néanmoins, je suis dubitatif quant à l'écart constaté et la récurrence du procédé. À mon sens, cela témoigne d'une volonté d'user d'un artifice comptable pour valoriser, en fin d'exercice, votre prétendue bonne gestion et pour valider de manière peu sincère votre théorie de la baisse d'impôt permanente. Pourtant, les temps que nous traversons nécessitent de la sincérité, préalable indispensable à l'obtention de notre confiance. Ce texte ne nous convainc pas ; c'est pourquoi le groupe SER s'abstiendra, du fait de mesures trop peu soucieuses de justice sociale.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour commencer mon propos, je veux emprunter à François-René de Chateaubriand l'une de ses fameuses maximes : « Presque toujours, en politique, le résultat est contraire à la prévision.

Il en résulte des dépenses en hausse de 70 milliards d'euros par rapport au budget initial, dont 3,8 milliards engagés dans ce projet de loi de finances aveugle à l'inflation galopante dans le pays ; vous en estimiez le taux à 1,5 % en décembre 2021, alors qu'il culmine à 5,3 % aujourd'hui. L'été venu, vous continuiez de le minorer de 0,3 Ce n'est pas uniquement le fait de la guerre en Ukraine, vous le savez : le bouclier énergie avait été instauré auparavant. Ce n'est pas uniquement le fait des difficultés d'approvisionnement, vous le savez : les producteurs et les distributeurs avaient déjà commencé à augmenter leurs prix.

Les aides sociales ont été revalorisées de 4 %, le point d'indice de 3,5 % : ces deux catégories de la population ont donc perdu du pouvoir d'achat. Dont acte ! Les travailleurs du secteur privé ont, eux aussi, vu fondre leur revenu au regard de l'inflation : on déplore 2,2 % de perte de pouvoir d'achat, en moyenne, pour les employés, 2,7 % pour les ouvriers, 3,6 % pour les professions intermédiaires et les cadres. Derrière ces moyennes, les ménages ne sont pas exposés de la même façon à l'augmentation de 11,2 % du prix des produits alimentaires sur l'année, ou à celle de 19,6 % du prix des produits énergétiques. Le travail ne paye pas suffisamment dans ce pays, donc l'État pallie, il tente de préserver un semblant de cohésion sociale. Lorsque le travail ne garantit pas les moyens de subsistance, c'est la Nation qui se délite. L'État sort donc son chéquier et tente d'alléger la facture. Tout y passe : l'électricité, les pellets de bois, les carburants, le fioul ... Plus de la moitié des crédits nouveaux ouverts par ce texte sont des palliatifs de l'envolée indécente des prix de l'énergie. La politique des chèques, c'est la politique des faibles La présidence française de l'Union européenne constituait pourtant une occasion de prendre des mesures structurelles pour soulager les peuples et les finances publiques : blocage du prix des carburants, en entamant des négociations serrées avec les producteurs et principaux exportateurs abrogation des directives de 1996 et 1998 de libéralisation du marché de l'énergie ; décorrélation des prix du gaz et de l'électricité. les finances publiques doivent assumer le coût de ces mesures. Vous procédez ainsi, monsieur le ministre, à plus de 6,8 milliards d'euros d'annulations de crédits ; surtout, vous nous resservez le discours d'une économie florissante, comme l'attesterait la hausse de 32,8 milliards d'euros des recettes fiscales par rapport à la loi de finances initiale.

par l'absence du partage de la valeur. Si l'économie se porte si bien, pourquoi donc la croissance, dont vous escomptiez au début de l'année qu'elle atteindrait 4 % du PIB, plafonne-t-elle à 2,7 % ? Le discours tenu autour du partage de la valeur m'incite à m'arrêter sur les 2 milliards d'euros alloués dans ce texte à France compétences. Je crois qu'il s'agit en vérité de « France patronat Ces 2 milliards d'euros ont pour seule vocation de subventionner l'emploi d'apprentis considérés comme une main-d'oeuvre à bon marché. L'apprentissage dans ces conditions de rémunération n'est pas une aubaine pour la France, c'est une aubaine pour le patronat

importantes. Du fait de cette absence de vision économique et budgétaire, du fait de l'absence de volonté de remédier structurellement aux maux provoqués par le libéralisme, si ce n'est par la politique des chèques, nous ne signerons pas en bas de la feuille, monsieur le ministre ! On ne signe pas un contrat lorsqu'il est défavorable aux intérêts les plus élémentaires de la population. Nous voterons donc contre ce texte, en vous donnant rendez-vous demain pour l'examen du projet de loi de finances

comme il est d'usage en fin d'année pour régulariser les crédits ouverts en fonction de prévisions plus proches de l'exécution réelle. C'est théoriquement le dernier texte de ce type.

Le texte présenté aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de ce paquet pouvoir d'achat, avec une rallonge de 2,5 milliards d'euros. C'est bienvenu, bien que cela s'inscrive dans un contexte budgétaire toujours Le Gouvernement propose 1,8 milliard d'euros pour financer un chèque énergie exceptionnel, prévoyant un versement de 100 ou de 200 euros qui sera effectué d'ici à la fin de l'année. Il aidera les 12 millions de ménages les plus fragiles à payer leurs factures énergétiques.

Dans la même logique, ce PLFR ouvre des crédits visant à couvrir les frais de carburant exceptionnels du ministère des armées, à hauteur de 200 millions d'euros ; 1,1 milliard

un million de foyers ! Il faudra que l'on y réfléchisse. La situation de l'économie française en cette fin d'année 2022 est certes incertaine, mais moins défavorable que celle d'autres pays.

En effet, si ce texte prévoit- et c'est heureux -un certain nombre d'aides ponctuelles sur lesquelles je reviendrai, il exprime aussi le dogme idéologique de la baisse de l'impôt et de la réduction de la dépense publique. Si la maîtrise de nos comptes publics est nécessaire, comme le souligne le Haut Conseil des finances publiques, disposer de marges de manoeuvre suffisantes pour faire face aux chocs macroéconomiques et aux besoins d'investissements publics ne peut se résumer à cette approche purement libérale, dont on mesure bien les limites et les dangers, et les dangers, singulièrement pour les plus modestes de nos concitoyens. Dans un contexte de crises multiples, vous avez fait le choix de verser des aides, qui sont tout de même de moins en moins exceptionnelles, pour soutenir le portefeuille des ménages. À défaut de politique structurelle, ce texte contient plusieurs mesures ponctuelles dont il convient de prendre acte favorablement face à l'urgence et aux difficultés de nos concitoyens.

afin que les étudiants puissent poursuivre leurs études dans des conditions acceptables. La nouvelle mouture des chèques énergies et l'aide à l'achat de carburant, même réduite, ne peuvent que contribuer à l'allégement des charges qui pèsent de plus en plus lourdement sur les ménages.

des réponses à apporter pour s'attaquer réellement aux inégalités sociales et revenir à un modèle de redistribution des richesses. À l'heure où la France compte 12 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, les mesures gouvernementales sont bienvenues, monsieur le ministre, mais elles ne sauraient vous exonérer de proposer des solutions pérennes permettant à nos concitoyens de vivre dignement. Pour ce faire, il est nécessaire d'en finir avec le désarmement fiscal et de conserver des recettes à la hauteur des enjeux. En cette fin d'exercice,

et si l'on peut remarquer que cette louable prudence s'est révélée un peu plus modérée qu'à l'accoutumée, ce supplément de recettes ne saurait trouver sa justification dans la baisse du taux de prélèvements obligatoires, comme l'avance le Gouvernement. Une baisse d'impôt est une baisse d'impôt : quelle que soit la manière dont on analyse les choses, ce sont bien des recettes en moins dans les caisses de l'État et, forcément, des recettes en moins pour le financement des politiques publiques et pour les services publics. Nous prenons donc acte, monsieur le ministre, des mesures d'urgence contenues dans ce texte et nous poursuivrons les débats, dans les jours qui viennent, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2023.

en août dernier, alors que nous entamions l'examen du premier projet de loi de finances rectificatives pour 2022, je m'étais inquiété devant vous du syndrome de « l'argent magique » et d'un « quoi qu'il en coûte » qui, étant dépourvu de bornes, l'était tout autant de sagesse Depuis lors, les taux d'intérêt, qui étaient restés négatifs et à peu près stables depuis 2019, n'ont cessé de poursuivre leur remontée. Sauf retournement, la prévision gouvernementale pour la fin de l'année 2022,

un coût annuel supplémentaire de 40 milliards d'euros pour le budget de l'État, soit l'équivalent du budget actuel de la défense. Mes chers collègues, la politique inconsidérée de dépense publique que permettait hier de financer sous anesthésie la Banque centrale européenne aura des conséquences très réelles, dont nous ne mesurons pas encore concrètement tous les effets négatifs quant à notre déclassement économique. de la première loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale, le déficit budgétaire de l'État tutoyait les 180 milliards d'euros, en hausse de près de 25 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Le second collectif budgétaire que nous ont transmis nos collègues députés affiche, du fait d'un grand nombre de crédits reportés, un solde qui s'améliore de plus de 5 milliards d'euros. Nous pourrions certes nous en réjouir. Le déficit budgétaire de l'État, dont on sait bien qu'il alimente une dette publique elle-même vertigineuse, reste cependant assez nettement supérieur à 170 milliards d'euros. Par égard pour les générations futures, nul ne peut vraiment

Beaucoup d'entre elles sont ciblées sur les publics les plus fragiles, par souci d'équité autant que de maîtrise des comptes publics. Le groupe Union Centriste, qui en appelle depuis le début de la crise à des mesures qui soient le plus justement calibrées, s'en réjouit. Mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt ! Nous ne pourrons pas éternellement dépenser sans compter et faire l'économie de réformes d'envergure. d'économies nouvelles et pérennes, afin de réduire significativement notre déficit et notre endettement publics, commanderait d'engager sans délai d'importantes réformes structurelles mise en oeuvre d'une réforme des retraites plus ambitieuse que celle qu'a annoncée le Président de la République ; réformes des prestations sociales et de l'assurance chômage ; réorganisation et redéfinition du périmètre de certains services publics, tels ceux de l'enseignement scolaire ou de l'audiovisuel, avec à la clef une baisse tangible tangible des effectifs ; report et même, dans certains cas, annulation des augmentations de crédits prévues dans le champ des politiques publiques non régaliennes ; et d'autres réformes encore. Plus tardifs seront nos efforts, plus brutal encore sera notre réveil ! La discussion

à M. le ministre délégué. Cet amendement vise à mettre à jour les prévisions sous-jacentes à ce projet de loi de finances rectificative pour 2022 concernant le déficit public et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l'article liminaire.

afin d'élargir la notion d'investissement initial aux biens de remplacement, la présente rédaction ne prévient en rien l'application restrictive déjà pratiquée par l'administration fiscale. nous craignons que la rédaction de cet article ne résolve pas le problème du financement des investissements de remplacement que nous souhaiterions éligibles au crédit d'impôt pour

monsieur le rapporteur

mondiale de la santé (OMS). L'accès à l'eau pour les besoins élémentaires est un droit fondamental. Or, alors qu'elle est pourtant indispensable à la vie, elle est facturée au même prix que l'eau destinée au remplissage des piscines ou à d'autres usages récréatifs. Ce n'est pas concevable. Il est essentiel que le prix de l'eau soit ajusté au besoin de tous et que cette denrée rare soit accessible en quantité suffisante. Tel n'est pas toujours le cas. En Guadeloupe, par exemple, un quart de la population n'a pas accès à l'eau au quotidien, du fait des nombreuses coupures, sans compter qu'on la paie beaucoup plus cher qu'en métropole. C'est dans cet esprit que le groupe Écologiste - Solidarité propose que les premiers mètres cubes d'eau soient exonérés de TVA. Cette franchise permettra une baisse de facture qui garantirait mieux le droit à l'eau dans la pratique. En outre, cet amendement s'inscrit dans la politique plus large que nous nous promouvons en faveur de l'accès à l'eau et aux énergies. Nous soutenons la multiplication des régies publiques, qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource et, souvent, une baisse de prix ainsi qu'une tarification sociale.

territoriales ont un rôle fondamental à jouer en matière de sécurité routière ; c'est pourquoi le projet de loi de finances prévoit d'ores et déjà les moyens adéquats issus des recettes de la police de circulation pour entretenir leur réseau et développer l'offre

son soutien indéfectible à l'investissement local au cours de ces dernières années, en particulier pendant la crise sanitaire et économique. Pour 2023, alors que le Gouvernement soutient les collectivités pour faire face aux conséquences de l'inflation par le filet de sécurité et l'abondement de la DGF- nous y reviendrons -, les crédits dédiés à l'investissement local sont également sanctuarisés, pour un montant total de près de 2 milliards d'euros.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

de 3,5 % du point d'indice, votée cette année, était donc essentielle, même si elle reste insuffisante, puisqu'elle ne couvre pas l'inflation de l'année en cours. Toutefois, les collectivités territoriales connaissent un contexte très défavorable, marqué par une inflation galopante, qui renchérit leurs dépenses de fonctionnement, et par la hausse exponentielle du coût de l'énergie.

Plus précisément, pour les communes dont la baisse d'épargne brute est comprise entre 20 % et 25 %, cet amendement tend à ouvrir droit à compensation d'une fraction réduite des dépenses d'approvisionnement, 35 % de la hausse des dépenses de personnel et 50 % de la hausse des dépenses d'énergie. En effet, une baisse arbitraire du seuil de 25 % conduirait à couvrir de la même manière des collectivités qui connaissent des situations financières pourtant très différentes et à reproduire ailleurs les effets de seuil du dispositif initial. À l'inverse, le mécanisme que nous proposons permettra d'apporter un soutien proportionné aux besoins réels des collectivités territoriales, d'en limiter le coût

que 20 000 communes puissent en bénéficier, car sans doute 20 000 en ont besoin.

augmentent de 907 ETP, ce qui porte à 1 942 377 le plafond des ETP. Cette augmentation concerne notamment le ministère de la justice- plus 605

les maisons France Services sont très majoritairement portées par les collectivités, surtout par les communes dans les quartiers prioritaires de la ville et plutôt par les intercommunalités en secteur rural,

de l'État, sachant que le coût moyen d'une maison France Services est d'environ 110 000 euros. De fait, il faut accompagner les collectivités qui se sont inscrites dans ce programme. Il s'agit, à travers cet amendement, de franchir une première marche,

L'idée est de renforcer et de soulager un peu les collectivités locales pour leur permettre de réorganiser le dispositif et, me semble-t-il, de trouver leur public, l'essentiel étant de permettre à tous les territoires, notamment aux territoires

à déployer encore davantage de partenariats au service des territoires. Il est important que l'État y prenne toute sa part. Nous sommes donc particulièrement favorables à cet amendement.

au Sénat, de proposer des dispositifs concrets, qui répondent à des besoins concrets, pour tout le territoire national.

de redéploiements et de remplacements de réseaux d'adduction dans les territoires. Cela a eu un vrai effet d'accélération-

écologiquement incontournable et porteur. Halte aux fuites ! Oui au soutien au déploiement du renouvellement des réseaux

Mme Sylvie Vermeillet. Tout comme les ménages chauffés au fioul et au bois, les 600 000 ménages chauffés au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ne disposent pas d'un accès au réseau de distribution de gaz naturel et ne bénéficient donc pas du bouclier tarifaire. Or le prix du propane, équivalent à celui du fioul, est près de 40 % plus élevé que celui du bois de chauffage. Aussi, en cohérence et par équité avec les dispositions votées pour les ménages se chauffant au fioul et au bois, le présent amendement vise à répliquer, à due proportion, le mécanisme d'aide pour les ménages se chauffant au propane. Quel

C'est un amendement pour finir à vingt et une heures, madame la présidente ... Les catastrophes climatiques s'enchaînent actuellement en France comme dans le reste du monde, et la dépendance aux énergies fossiles pose un problème dont chacun a désormais conscience. Le Gouvernement a annoncé des mesures de sobriété destinées à limiter les effets de l'inflation et de notre dépendance aux fossiles. Le passage à 110 kilomètres par heure que nous vous proposons est une mesure efficace, immédiatement applicable, très simple à mettre en oeuvre, très peu coûteuse pour l'État, profitable aux automobilistes. Elle avait, de surcroît, je le rappelle, était proposée par la Convention citoyenne pour le climat.

énorme en termes d'économies de carburant- d'environ 20 % - et de réduction des gaz à effet de serre- d'environ 25 %. Elle nous permettrait, en outre, d'être moins dépendants aux énergies fossiles et d'améliorer notre balance au commerce extérieur. La gravité de la situation écologique justifie de telles mesures,

Cet amendement vise à prévoir une nouvelle dotation pour permettre de réaliser les travaux d'insonorisation chez les riverains des grands aéroports. Le transport aérien

devons verser ces droits de douane en 2022.

Notre collègue Michel Canévet a parfaitement résumé l'état d'esprit de beaucoup de sénatrices et de sénateurs quant à la poursuite de la création d'emplois

à ces créations de postes, qui représentent un solde net supplémentaire. Vous partagez parfois avec notre assemblée la volonté de maîtriser la dépense publique. Les auteurs de cet amendement vous y invitent.

doublement du déficit foncier déjà permis dans la limite de 10 700 euros ne doit pas exonérer d'effort financier les bailleurs privés dans la réalisation des travaux de rénovation

L'association Attac a développé l'exemple suivant : un célibataire qui déclare 30 000 euros de salaire pour seuls revenus au titre de 2021 aura payé 2 022 euros d'impôts en 2022. Les choses sont bien faites : si l'on prend son barème, le taux marginal appliqué à son revenu sur sa dernière tranche est de 30 %. qui l'informe réellement ? Non, car son taux réel d'imposition est de 6,74 %. Cet exemple, aussi beau soit-il, concerne un célibataire sans autres revenus que son salaire. Si l'on ajoute à cela le bénéfice d'une ou plusieurs des 180 niches fiscales à l'impôt sur le revenu, la lisibilité du taux moyen est largement altérée.

pourquoi nous proposons l'instauration d'une véritable progressivité de l'impôt sur le revenu grâce à onze tranches. Vous vous y opposez systématiquement.

Cela créerait un sentiment partagé et concret d'attachement à nos services publics. Ce que l'on paye par l'impôt, on ne le paye pas à la caisse ! C'est trivial, mais c'est factuel.

d'autant que les dispositifs proposés semblent raisonnables et s'inspirent de ce qui s'est déjà fait en matière d'éolien. Je rappelle par ailleurs que cet article est le fruit d'un consensus trouvé à l'Assemblée nationale, au-delà des clivages.

à une délibération en conseil municipal. Celui-ci n'a donc rien d'automatique et ne remet pas en question les équilibres existants. Nous vantons souvent ici les mérites de la proximité. Il me paraîtrait illogique

Le partage de la valeur doit se faire à l'échelle du territoire investi par les énergies renouvelables (ENR). Pour le développement du photovoltaïque, c'est bien à l'échelle des communes d'implantation que l'acceptabilité doit être

ce n'est pas une solution. Cela reviendrait en quelque sorte à mettre en concurrence les collectivités les unes avec les autres en niant le rôle des départements dans l'implantation d'installations photovoltaïques,

les EPCI à fiscalité additionnelle, qui sont avantagés par la procédure actuelle, des EPCI à fiscalité professionnelle unique,

Depuis la loi de finances pour 2022, les communes qui instaurent la taxe d'aménagement ont l'obligation d'en reverser tout ou partie à l'intercommunalité. Nous considérons que cette obligation est inutile, contraignante et source de conflits. Le groupe

Nous souhaitons revenir à la situation qui prévalait avant la loi de finances pour 2022, ce que ne permet pas l'amendement que vous avez fait adopter dans le PLF.

amendement est en partie contraire à l'objectif du Gouvernement d'accélérer la production d'énergies renouvelables, dans la mesure où le dispositif proposé majorerait la valeur forfaitaire de la taxe d'aménagement appliquée aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques, alors qu'ils contribuent au développement d'une énergie renouvelable et durable.

En application de l'article 47 , alinéa 3, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une coordination de l'article d'équilibre, article 3 et état A, du projet de loi de finances rectificative pour 2022. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de coordination ? Avis favorable.